L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement

Actuellement, lors d'une perquisition, alors que le mis en cause a signé l'assentiment, il peut décider de quitter les lieux. L'investigation s'arrête alors. Le seul moyen de le contraindre est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue, limitée dans le temps, de six heures permettrait de poursuivre et de terminer la perquisition. Il est dès lors proposé, afin de renforcer l'action de la police de l'environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d'introduire un article L. 172-8-1 dans le code de l'environnement créant une retenue environnementale inspirée de la retenue douanière.

qui ferait suite à une arrestation prononcée par un inspecteur de l'environnement. Il s'agit d'une attribution manifeste d'une prérogative exclusivement exercée par un OPJ, et qui s'apparente, hormis les délais, à une forme de garde à vue. En cohérence

Une retenue requiert des locaux adaptés, ainsi qu'une expérience avérée de gestion des personnes placées sous une telle contrainte que seule une pratique régulière permet d'acquérir. En cas de nécessité, l'article 47 de la loi Justice, qui vient d'être promulguée, facilitera les cosaisines avec un officier de police judiciaire. L'avis

Ces trois amendements ont donc pour objet de renforcer les pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement en accroissant notamment leurs pouvoirs d'investigation et en leur attribuant, sous des conditions précises et encadrées par le juge des libertés et la possibilité d'intercepter des communications électroniques ou téléphoniques, ce qui est très utile en cas de braconnage et de trafic animalier.

tend à étendre aux inspecteurs de l'environnement la capacité réservée aux officiers et agents de police judiciaire de mettre en oeuvre la procédure applicable en cas de crimes ou de délits commis en bande organisée portant atteinte au patrimoine naturel. Là encore, compte tenu du nombre, des moyens et de la formation des inspecteurs de l'environnement, cet amendement paraît quelque peu disproportionné, mais surtout peu compatible avec les réalités de terrain. J'en profite pour indiquer

pour la recherche d'individus soupçonnés d'actes de terrorisme, de meurtre ou de tout autre délit ou crime puni d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Il a semblé à la commission que cette disposition était quelque peu disproportionnée. En conclusion, l'avis de

Nous avons travaillé dans deux directions : premièrement, le projet de loi a déjà augmenté significativement les pouvoirs des officiers de police de l'environnement en matière de réquisition, de saisine, d'accès aux fichiers de la justice et de la police ; deuxièmement, dans le cadre de la loi Justice, qui vient d'être

est à M. Jérôme Bignon. En 2018 a été instaurée l'obligation pour les inspecteurs de l'environnement de transmettre systématiquement une copie du procès-verbal de constatation aux contrevenants, sauf si le procureur de la République ne le souhaite pas.

Préville, pour présenter l'amendement n° 142. L'ordonnance d'harmonisation des polices de l'environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux qui appartiennent à la fonction publique, territoriale ou d'État. En effet, les seconds disposent de l'ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l'environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu'une partie. Cela est particulièrement regrettable lorsque l'on sait que 55 l'on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs. Conformément à l'article R. 332-20 du code de l'environnement, « le gestionnaire de la au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. » À cette fin, l'agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Cet amendement n'a pas pour objet d'octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d'une mission de service public l'ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, mais il vise à renforcer les pouvoirs des premiers s'agissant de la communication entre agents d'informations et de documents recueillis dans l'exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de la destruction après saisie des végétaux et animaux morts non viables ou bien du prélèvement d'échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Cela permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles. J'insiste sur deux points.

ne s'agit pas de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agent public. Cependant, en leur accordant quelques moyens d'action supplémentaires, on pourrait renforcer grandement leur capacité d'action.

En cohérence avec la position qu'elle a adoptée au moment de l'examen du texte en son sein en faveur de l'extension des compétences de police des agents des réserves naturelles, la commission verrait d'un oeil favorable

: il vise à étendre le domaine d'intervention des agents spécialisés des fédérations des chasseurs dans le cadre de l'application des schémas départementaux de gestion cynégétique,

au constat par procès-verbal et à la seule aire géographique couverte par la fédération. La rédaction ainsi proposée pourrait convenir si les compétences des agents des fédérations étaient calquées sur celles des gardes particuliers assermentés,

parole est à Mme Michèle Vullien. L'affectation à titre gratuit de biens saisis ne doit être possible que pour les services de police, les unités de gendarmerie ou l'administration des douanes. Le futur office français de la biodiversité et de la chasse ne saurait jouir des mêmes possibilités,

pour ces agents de l'office entre le statut d'officier de police judiciaire et la capacité à disposer des meilleurs moyens pour mener leurs enquêtes. Sur ce point particulier, l'affectation de biens saisis correspond à un réel besoin et il n'y a pas de raison de les traiter différemment des membres de la police, de la gendarmerie et des douanes. Madame

Ainsi, comme le souligne la loi de 2005 relative à l'aménagement rural, celui-ci a pour but de répondre aux attentes de tous les acteurs du monde rural et concerne, au même niveau, l'agriculture, l'environnement et l'aménagement du territoire, dans une logique de développement durable. Il doit contribuer, depuis 2010, à préserver la ressource en eau, la biodiversité et les continuités écologiques entre les milieux. Nature Environnement, ces opérations lourdes d'aménagement, qui tendent les rapports aux paysages pour des motifs d'échanges de propriété, s'accompagnent traditionnellement d'importantes atteintes à la biodiversité, qui justifient le régime de protection conservatoire mis en place par le législateur depuis 1993.

ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement ». C'est pourquoi nous proposons que tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel puissent exercer les pouvoirs de police dévolus aux seuls agents des services de l'État ou des conseils départementaux.

Le Gouvernement ne souhaite pas renforcer les moyens de l'État ou de ses établissements sur cette mission décentralisée. Par ailleurs, l'élargissement du nombre d'agents habilités n'apporterait pas de garantie quant à l'effectivité des contrôles, car les agents de l'office ne disposent pas, à ce stade, de compétences techniques associées.

le conseil aux administrations et l'expertise scientifique, l'AFB avait initialement pour mission de mobiliser la société civile et de créer des liens entre les acteurs de la défense de l'environnement et la population française.

et, dans l'esprit de l'AFB, de développer le lien entre l'État et les citoyens. Il s'agira d'un véritable trait d'union, utile pour les missions de police, mais aussi pour les conseils techniques que pourraient apporter de nombreux réservistes à l'institution. Ainsi, de nombreux agents partant à la retraite auraient la possibilité de continuer à servir l'État. Il est même prévu une indemnisation que le Gouvernement pourrait adapter. Cet amendement s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle ; il est porteur d'une vision optimiste et participative et vise à renforcer le lien entre l'État et la société civile.

Ainsi, le Comité national de la conchyliculture nous a fait parvenir plusieurs exemples dans lesquels les comités régionaux des pêches et, surtout, les comités de la conchyliculture s'étaient vus refuser le droit de se constituer partie civile au motif que l'infraction était relative à la protection de la nature et de l'environnement, prévue au code de l'environnement. Pourtant, la participation aux politiques publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement est une mission légale qui incombe aux comités des pêches. De la même façon, les comités de la conchyliculture sont chargés de missions de service public ; ils doivent, notamment, participer à la protection, à la conservation et à la gestion des milieux

L'amendement qui vient d'être présenté a pour objet de permettre aux comités des pêches et de la conchyliculture d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'une infraction environnementale.

toutes les capacités d'être reconnu en tant que partie civile face à des infractions, quel que soit le code retenu. Le Gouvernement vous soumet donc le sous-amendement n° 218, qui tend à inscrire cette compétence dans le code rural et de la pêche maritime.

ou un ouvrage après cessation d'activité. En effet, aucune peine n'est aujourd'hui prévue s'agissant des installations et des ouvrages qui ne sont plus exploités et qui doivent être remis en état, conformément à la législation.

portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et, en l'espèce, renforçant la police de l'environnement. Il tend à expliciter dans le code de procédure pénale que les inspecteurs de l'environnement sont constitués en service de police judiciaire pour l'exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, leur permettant ainsi de bénéficier de tous textes faisant référence aux services de police. Ils auront notamment la possibilité d'utiliser des avertisseurs spéciaux, tels que gyrophares et sirènes hurlantes, et de bénéficier des biens qu'ils

Les problèmes de hiérarchisation judiciaire et de résolution des enquêtes trop complexes seront résorbés par ce service qui permettra un meilleur traitement du renseignement. La délinquance environnementale sera mieux identifiée et combattue à la possibilité de mettre en oeuvre tous les moyens prévus dans le code de procédure pénale. La police de l'environnement bénéficiera ainsi de nouveaux moyens de coercition, sous l'autorité d'un magistrat, notamment les auditions sous contrainte, les perquisitions sans assentiment et les mesures d'enquête telles que les écoutes ou la géolocalisation.

en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l'OFBC des prérogatives similaires à celles qui sont consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux, en leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des OPJ lorsqu'ils sont requis par l'autorité judiciaire en la personne du procureur de la République ou d'un juge d'instruction.

entre les inspecteurs de l'environnement et ceux qui, en fonction de leurs compétences et de leur appétence, pourraient être amenés à devenir des officiers judiciaires de l'environnement. Quel est l'avis de la commission ?

prévoit notamment la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement d'être requis par le procureur de la République ou par commission rogatoire du juge d'instruction : cette disposition est satisfaite par le texte de la commission.

La commission entend que le périmètre de compétence des inspecteurs de l'environnement et des autres fonctionnaires et agents publics de police environnementale soit étendu à un socle commun d'infractions. Elle est donc défavorable à ces deux amendements. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis pour les deux amendements.

a été au rendez-vous. Face à cette problématique, c'est le maire qui est désigné responsable par la réglementation, quand bien même elle le dote de peu de moyens de contrainte.

afin de le mettre en demeure d'enlever les déchets. Dans les faits, compte tenu de ses responsabilités, vous vous doutez bien que le maire fait enlever les déchets par ses services, quand il en a. En la matière, très clairement, l'absence de sanction fait perdurer le geste.

la vidéoprotection à des fins de prévention permet déjà d'inclure le recueil de preuves pour la répression d'infractions en matière d'abandon de déchets. Vous savez combien les chasseurs sont vigilants et respectueux de l'environnement et de la biodiversité en général, notamment quand il s'agit de déclarer des abandons de déchets. proposée de la verbalisation ne serait pas opportune, car la vidéoverbalisation qui pourrait être mise en place avec un dispositif de verbalisation automatique poserait de sérieux problèmes de constitutionnalité. on ne peut pas établir de lien direct et systématique entre la propriété d'un véhicule et la commission d'une infraction en matière d'abandon de déchets : certains particuliers pourraient se voir sanctionnés

un producteur de déchets de se mettre en conformité avec la réglementation en la matière., un dispositif se fondant sur des notions de droit pénal,

évidemment, nos maires ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on leur fournisse les moyens d'entretenir et de conserver les biens dont ils sont garants. Donnons-leur des outils simples ! On ne parle pas forcément de l'entreprise qui se débarrasse d'un camion entier de déchets, mais plutôt du manque

monsieur le rapporteur,

de montrer que vous avez écouté le grand débat. Pourquoi ? Nos collègues se sont exprimés, par-delà la diversité ; ce sujet est un fléau un fléau dans notre pays, que l'on soit maire de commune rurale, péri-urbaine ou urbaine. Plutôt que d'opposer une réponse technique à un problème concret et pratique,

conduite par M. Ettore Licheri, président de la commission des affaires européennes. Nos collègues italiens ont eu ce matin une réunion conjointe avec notre commission des affaires européennes, qui se poursuivra tout à l'heure autour d'un déjeuner de travail. L'accueil de cette délégation, quelques mois après que nos collègues ont été reçus à Rome, est l'occasion de poursuivre un dialogue ininterrompu entre nos commissions des affaires européennes. Au nom du Sénat de la République, je souhaite la plus cordiale bienvenue à nos collègues italiens et je forme des voeux pour que leur séjour en France leur soit profitable et permette de renforcer les liens qui unissent nos deux pays. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 500 anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, puisse-t-il inspirer nos prochains pas et nous guider dans le développement pluriséculaire de l'amitié entre l'Italie et la France, à laquelle le Sénat de la République française est foncièrement attaché. je vous remercie

parole est à Mme Sylviane Noël. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié le quantum des peines requis pour l'emploi de moyens nécessaires lors de la phase d'instruction. Le minimum des peines délictuelles pour déployer ces moyens est désormais de trois ans d'emprisonnement. Par conséquent, pour enquêter sur commission rogatoire pour démanteler les réseaux de trafiquants de spécimens d'espèces de faune ou de flore sauvages menacées d'extinction ou de gibiers, il est proposé de mettre en cohérence le quantum des peines d'emprisonnement prévu par cette réforme avec celui qui est fixé par le code de l'environnement pour les peines concernant les atteintes aux espèces protégées et le braconnage. Cette réforme pour la justice comporte également une révision du code des douanes, ramenant de cinq à trois ans le quantum de la peine d'emprisonnement nécessaire à la mise en oeuvre de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes douanières.

peuvent recourir à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel pour tout auteur de crime ou de délit punissable d'une peine d'emprisonnement de trois ans à trois ans la peine applicable aux crimes et délits allant à l'encontre de la conservation et de la protection des espèces animales et végétales, cet amendement permet de faire en sorte que le dispositif de géolocalisation évoqué, dont je rappelle qu'il ne sera ouvert qu'aux seuls OPJ, leur soit appliqué.

À l'intérieur de ces parcs, certains biens ont été choisis par la France pour être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le cas, par exemple, du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui possède en son sein la chaîne des Puys, proposée par la France et inscrite au patrimoine de l'Unesco l'an dernier. Cette inscription repose également sur une obligation de préservation et de conciliation des usages. Or, aujourd'hui, les gardes nature des parcs régionaux ne peuvent pas assurer correctement leur mission puisqu'ils sont toujours dans l'attente d'un décret, dont la rédaction est sans cesse repoussée depuis l'adoption de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L'objet de cet amendement est d'inciter le Gouvernement à publier ce décret au plus vite avant la période estivale, qui verra naturellement le nombre de visiteurs augmenter dans les parcs naturels régionaux. Il est essentiel de permettre à ces agents, au-delà de leur mission de prévention et d'information, de rechercher et constater les infractions pour assurer une protection efficace de notre patrimoine naturel. Quel

a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administratives de ce permis uniquement en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse. de chasse. Le 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant soixante-douze heures à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat d'incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui. Cette rétention est aussi prévue en cas d'accident au cours d'une action de chasse ou de destruction ayant causé un homicide involontaire ou une atteinte involontaire et grave à l'intégrité de la personne. la personne. Le 2° définit les sanctions judiciaires en cas de non-respect des mesures de rétention ou de suspension administratives du permis de chasser. Il élargit par ailleurs le champ de la peine judiciaire complémentaire de suspension de ce permis aux cas où aurait été constatée une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Il s'agit de réagir aux cas dans lesquels

accidentellement une voiture dans laquelle se trouvaient trois enfants. La balle a brisé la lunette arrière et s'est logée dans le coffre du véhicule. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, donc pas

entre les services et avec bon nombre de collègues ici présents. Vous avez rappelé l'accident qui a eu lieu dans le Gers, accident qui aurait pu être dramatique, nous en convenons.

sens d'une meilleure responsabilisation collective de la chasse et des pratiques de chasse vont dans le bon sens et permettent une meilleure transparence de ces pratiques et, sans doute, une meilleure compréhension. En l'espèce, cet amendement constitue une avancée, et nous le soutenons. La

-, qui vont jusqu'à des attaques à l'intégrité des personnes et des animaux. Certains antispécistes perturbent les chasses à courre ; ils ont provoqué la chute, en Bretagne, d'un homme de vénerie à cheval qui a eu deux membres fracturés et est resté des mois à à l'hôpital. Parallèlement, ces mêmes personnes tentent d'empoisonner les chiens qui chassent. On peut être antichasse et plaider en faveur des animaux, mais il faut mettre ses actes en corrélation avec ce que l'on préconise. Je le

chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de dire qu'il n'est pas d'accord, mais personne n'a le droit d'empêcher quiconque par la force et la violence d'exercer une activité légalement autorisée. La parole est

Le reclassement en délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents chargés de la police de la chasse, ainsi qu'aux forces de l'ordre, d'intervenir pour sanctionner les auteurs d'obstructions violentes dont sont victimes les chasseurs. La répression de l'acte d'obstruction à un acte de chasse, considéré comme un délit, suppose d'adopter un texte de loi, conformément à l'article 111-3 du code pénal, et de supprimer par décret en Conseil d'État l'article R. 428-12-1 du code de l'environnement.

Gouvernement ? Monsieur le sénateur Cardoux, vous avez déposé le 9 octobre dernier une excellente proposition de loi tendant à réprimer les entraves à l'exercice des libertés ainsi qu'à la tenue des événements et à l'exercice d'activités autorisés par la loi. Elle pose la question de savoir comment on peut créer un délit d'entrave sur toutes les activités légales, qui doivent pouvoir être exercées de façon paisible dans ce pays et qui, pour une raison ou une autre, font l'objet d'entraves. Je soutiens l'inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour des assemblées, parce que je pense qu'il est de nature à permettre de traiter la question que vous posez aujourd'hui. La chasse est évidemment une activité légale qui doit pouvoir être exercée en toute tranquillité, mais il me semble que le sujet, qui soulève une question juridique importante, peut et doit être traité de façon transversale. En attendant, une contravention de cinquième classe d'obstruction à la chasse existe déjà ; elle sanctionne à hauteur de 1 500 euros d'amende- montant qui peut être doublé en cas de récidive, soit 3 000 euros d'amende -les actes d'obstruction les plus graves. Les faits que vous avez mentionnés, qui sont évidemment répréhensibles, peuvent être poursuivis selon des incriminations de droit commun, dès lors qu'il y a violence physique ou même en cas de menace. Le passage d'une contravention à un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut présenter un intérêt procédural, mais peut aussi être considéré comme disproportionné.

de loi à votre compte, puisque vous venez de nous dire qu'elle était excellente. Mettez une fois pour toutes vos paroles en conformité avec vos actes

celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

En pleine complémentarité avec les inspecteurs de l'environnement, ils assurent une police de proximité, sans avoir pour autant vocation à assurer une police de nuit avec des armes de service.

Ce projet de loi fait l'impasse sur ce sujet en reléguant cette dépense aux seuls forestiers. Il s'agit là, nous le savons, d'une ligne rouge, les chasseurs mettant en avant leur incapacité à assumer de telles charges supplémentaires. Certes, mais le sujet existe bel et bien : si les seuls forestiers doivent désormais assurer ces surcoûts grandissants, il convient de les associer étroitement, et dans un esprit de responsabilisation, à l'élaboration des plans de chasse.

relevé Jean-Noël Cardoux dans le cadre de sa mission sur les dégâts de grand gibier, une telle évolution impliquerait des besoins de financement supplémentaires considérables, appelant une ressource spécifique

instaure déjà un dispositif d'indemnisation à la charge du bénéficiaire du droit de chasse. Par ailleurs, je renvoie également au rapport de MM. Cardoux et Perea sur les dégâts de grand gibier, qui précise que les indemnisations des dégâts forestiers ne sont envisageables qu'en cas de nouvelle source de financement dédiée. La parole est à M.

: le dialogue entre forestiers et chasseurs est extrêmement étroit et efficace, et a produit des résultats très fiables. En revanche, nous avons tout de même ouvert une petite porte dans notre rapport, après avoir entendu les forestiers.

Le fonds alimenté par les fédérations à partir du prélèvement minimum de 5 euros par chasseur, que le type de validation soit départemental ou national, doit être géré par la

de loi prévoit, entre autres mesures, l'instauration d'une obligation, pour la Fédération nationale et les fédérations départementales des chasseurs, de mener des actions concourant à la protection de la biodiversité, en y consacrant un minimum de 5 euros par chasseur à l'échelon départemental et national. L'État, pour sa part, à la suite d'une promesse du Président de la République, y participera à hauteur de 10 euros par chasseur. Comme cela a été rappelé, le Gouvernement est incapable de répondre sur la manière dont il entend financer cette contribution, ce qui porte en germe le risque d'un nouveau prélèvement sur le budget des agences de l'eau, déjà sérieusement ponctionné par ailleurs. En outre, de nombreuses questions demeurent s'agissant de la mise en oeuvre desdites actions. On a évoqué une convention-cadre entre les fédérations et l'État, un fonds national et, plus récemment, des appels à projets, dont les modalités restent à préciser. Dès lors, tant que le flou persiste sur cette contribution, nous souhaitons revenir sur son inscription, par la commission de l'aménagement du territoire

les fédérations départementales financeront des actions à hauteur de 5 euros par adhérent ayant un permis départemental et, de ce fait, recevront par convention un soutien de l'État à hauteur de 10 euros par adhérent d'autre part, la Fédération nationale des chasseurs gérera un fonds alimenté par sa contribution fixée à 5 euros par permis national, ainsi que par une contribution de l'État à hauteur de 10 euros par permis national. L'objectif est le suivant : chaque fédération départementale recevra une juste contribution de l'État, au regard de son nombre d'adhérents et des efforts qu'elle va réaliser, et le fonds géré par la FNC assurera une péréquation complémentaire entre fédérations départementales. L'amendement proposé tend à centraliser l'ensemble des financements dans le fonds géré par la FNC,

l'amendement n° 164 revient sur un apport important de la commission. Il s'agit de graver dans la loi l'engagement pris par le Gouvernement de contribuer à hauteur de 10 euros par permis

Une telle mesure aurait pour conséquence d'alourdir excessivement le dispositif, en conférant à une structure un droit de regard considérable sur l'utilisation des ressources des fédérations départementales des chasseurs. Cet amendement me semble satisfait par l'introduction, en commission, d'une convention entre l'État et chaque fédération, qui impliquera nécessairement l'OFBC, représentant les acteurs agro-sylvo-cynégétiques, et permettra de préciser les actions éligibles au financement public. En outre, comme cela se fait déjà, des partenaires publics et privés, notamment agricoles et forestiers, contribueront aux actions des fédérations, avec, nécessairement, un dialogue entre les parties prenantes.

M. Jean-Paul Prince. Le présent amendement vise à améliorer la rédaction du texte de la commission en vue de confier aux fédérations des chasseurs une responsabilité générale de collecte et de production de données.

présent amendement tend donc à consacrer cette responsabilité et à définir les principes de transmission des données ainsi recueillies à l'office français de la biodiversité et de la chasse. Quel est l'avis de la commission ?

à la demande de ce dernier, gratuitement et sans délai. Supprimer le principe d'une transmission à la demande risque de faire peser une contrainte excessive sur les fédérations, sachant, par ailleurs, que plusieurs dispositifs spécifiques de transmission de données précisent le rythme ou l'initiative des transmissions, notamment pour le fichier central des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser ou les données de prélèvement sur la gestion adaptative. La commission émet donc un avis défavorable.